J'informe le Sénat que la commission mixte paritaire chargée d'élaborer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi confortant les principes de la République et de lutte contre le séparatisme n'est pas parvenue à l'adoption d'un texte commun. texte commun. Par lettre en date du 12 mai 2021, M. Guillaume Gontard, président du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires, a demandé l'interversion des textes inscrits à l'ordre du jour de l'espace réservé à son groupe du mercredi 26 mai En conséquence, la proposition de loi d'urgence visant à apporter une réponse solidaire et juste face à la crise sera examinée avant la proposition de loi pour un élevage éthique, juste socialement et soucieux du bien-être animal. Acte est donné de cette demande.

européen, sans droits de douane et sans quota, d'un certain nombre de produits au respect d'une quinzaine de conventions internationales, dont plus de la moitié sont des conventions de l'Organisation internationale du travail (OIT). Loin d'être des gadgets, ces clauses donnent un poids beaucoup plus

Mme Jacky Deromedi. Cet amendement a pour objet de faire concrètement de la commande publique et de l'aide au développement de véritables leviers de développement durable et de renforcer la dynamique vertueuse des critères de responsabilité sociétale des entreprises

universellement acceptés, touchant les droits de l'homme, les normes du travail, l'environnement et la lutte contre la corruption. Ces critères permettront également de considérer un marché en fonction de son coût global et non plus du coût initial des fournitures et des travaux. Les enjeux de durabilité, de cycle de vie des produits et de coût de la maintenance doivent être aussi pris en compte, comme le précise le rapport annexé au projet de loi au sujet de « l'assistance technique cruciale » que la France doit apporter « pour garantir la durabilité des produits concernés par les différents projets

De nombreux pays, qui ne respectent pas les mêmes standards que les pays européens en matière sociale et environnementale, développent leurs industries grâce aux marchés publics financés par l'aide au développement française. La commande publique et l'aide au développement doivent devenir de véritables leviers de développement durable et enclencher une dynamique vertueuse en matière de responsabilité sociale et environnementale. Il semble dès lors nécessaire d'inscrire la commande publique dans les enjeux contemporains, en soutenant l'harmonisation des normes de entre les États, tout en préservant les intérêts de la France. Dans ce but, le présent amendement vise à favoriser- là est la différence avec les autres amendements -la prise en compte des critères sociaux et environnementaux dans les clauses des marchés publics financés par l'aide au développement française et, le cas échéant, à les renforcer pour les marchés publics qui en sont déjà dotés.

et environnementale, notamment la défense de l'environnement, le respect du droit du travail et des droits syndicaux, l'interdiction du travail forcé, la non-corruption ainsi que les droits de l'homme. Il s'agit d'encourager ainsi les entreprises soumissionnaires aux marchés à mieux respecter les valeurs qui sont en phase avec les principes de l'aide au développement, à l'image des critères du Pacte mondial des Nations unies et de ses dix principes universellement acceptés, touchant les droits de l'homme, les normes du travail, l'environnement et la lutte contre la corruption. À l'heure où « notre maison brûle », pour reprendre les mots du président Chirac, cette mesure permettra de faire concrètement de la commande publique et de l'aide au développement de véritables leviers de développement durable.

La promotion de la RSE et les critères de durabilité, mais également la lutte contre la concurrence déloyale, sont des thèmes sur lesquels nous pouvons tous nous rejoindre. Toutefois, il paraît difficile d'imposer aux pays partenaires ces exigences dans leurs propres marchés publics, même dans le cadre de projets financés par l'AFD ou par le ministère des affaires étrangères.

effet, elle est très incitative, elle s'inscrit bien dans les priorités françaises et européennes et elle vise à renforcer la dimension sociale et environnementale des activités de l'aide au commerce. En revanche, elle n'est pas prescriptive

Il tend à réserver l'accès aux marchés publics de l'aide au développement aux entreprises originaires des pays bénéficiaires de cette aide et aux entreprises des pays parties à l'accord sur les marchés publics de l'Organisation mondiale du commerce

Le France, dans le cadre de sa diplomatie féministe, doit promouvoir l'égalité entre les femmes et les hommes à tous les échelons. L'adoption de cet amendement permettrait d'affirmer la conception forte de l'État de droit que la France se doit de porter dans le cadre de son aide publique au développement

L'alinéa 104 du CPG fixe les objectifs que la France promeut dans les politiques de développement urbain, en particulier en Afrique : « l'accès aux services essentiels, l'attractivité et la prospérité des territoires ou encore la protection de la santé des citoyens et de l'environnement Y ajouter l'accès à la pratique sportive est important, tant l'activité physique est un facteur essentiel de santé, en particulier dans un contexte urbain où la sédentarité des modes de vie s'accroît. unies consiste à « faire en sorte que les villes et les établissements humains soient ouverts à tous, sûrs, résilients et durables ». Le Comité international olympique (CIO) s'est engagé en faveur de cet objectif, soulignant que « les villes qui investissent dans des terrains de sport et des espaces de jeu publics ainsi que dans des programmes d'activités physiques et sportives parviennent à économiser de l'argent sur les soins de santé, à lutter contre la délinquance et la violence, et à promouvoir la cohésion sociale et l'identité communautaire. Les évènements sportifs peuvent également permettre d'accélérer le développement de villes durables, notamment avec des réseaux routiers et des transports publics améliorés, contribuant ainsi à la sécurité routière ». De nombreux acteurs engagés dans la politique de développement sont conscients de l'importance du sport et leurs axes d'action se renforcent fortement autour de cette problématique. C'est pourquoi cet amendement tend à mentionner spécifiquement l'apport du sport et de la pratique des activités physiques et sportives dans le cadre de la mise en place des politiques urbaines. Quel est l'avis de de la commission ? Nous avons été très attentifs à la thématique sportive depuis le début de cette discussion. Toutefois, la mention de la pratique sportive ne paraît pas indispensable dans un alinéa qui cite comme grands axes de la politique de développement solidaire, en relation avec le fait urbain, « l'inclusion sociale, l'accès aux services essentiels, l'attractivité et la prospérité des territoires ou encore la protection de la santé des citoyens et de l'environnement ». La commission a donc émis un avis défavorable

et du microcrédit dans les pays partenaires. Elle accompagne le déploiement à l'international des acteurs de l'ESS et renforce les initiatives locales en favorisant l'accès aux financements et la structuration d'écosystèmes. » Cela nous semble suffisant et de nature à satisfaire cet amendement.

amplifier la lutte contre les paradis fiscaux, qui, au-delà de leur immoralité, participent à l'aggravation des inégalités en captant les fonds destinés aux services de base.

commission ? La lutte contre l'évasion fiscale est mentionnée aux alinéas 105 et 144 du CPG, aux termes desquels la France s'engage dans la lutte contre l'évasion fiscale, l'opacité financière et les flux financiers illicites.

libellé : La parole est à M. André Gattolin. La question du développement de l'économie numérique et des installations numériques est stratégique pour l'ensemble de la planète, en particulier pour les pays en développement. Aussi, cet amendement tend à appeler la France à soutenir une politique de développement dédiée politique de développement dédiée à la réduction de la fracture numérique, à l'accompagnement de la révolution numérique dans les pays en développement et à la mobilisation de nouvelles technologies pour la réalisation du fameux Agenda 2030, dont plus spécifiquement les cibles de l'ODD 9. Dans ce cadre, il est important que notre politique de développement contribue au développement d'infrastructures critiques,

Dans le cadre de ses relations internationales, l'État français veille au respect de la souveraineté des États. À ce titre, cet amendement tend à prévoir, en plus de la possibilité initialement prévue de restitution des recettes issues de la cession des biens confisqués, la possibilité d'une restitution des biens eux-mêmes lorsque ceux-ci sont susceptibles de participer à l'action diplomatique de l'État concerné. Ainsi, les modalités et l'objet de la restitution seraient appréciés au cas par cas, afin de permettre une restitution adaptée aux besoins de l'État concerné et d'éviter la cession d'un bien qui pourrait profiter à l'action diplomatique de l'État concerné. Quel est l'avis de

le Premier ministre est contraint de le réunir au moins une fois par an. Quel

la politique nationale ne convient pas. Elle consiste précisément à renforcer une dérive institutionnelle qui est à la source de beaucoup de problèmes quant à la mobilisation citoyenne de la société. Puisque vous parlez des ONG, il y aurait bien d'autres choses à faire pour donner plus de place à la société civile que de donner des pouvoirs

Carlotti. Le projet de loi instaure un triple pilotage de la politique de développement par le ministre chargé du développement, le ministre du budget et le ministre de l'économie. On sait que la pression de Bercy est toujours très forte, mais, en l'occurrence, on peut y voir sa tutelle. Si l'ambition de la France est de renforcer sa politique de développement, si l'ambition du Gouvernement est de clarifier sa politique au regard des Français, si l'on veut un suivi et un accompagnement permanents d'une politique de plus en plus complexe et mondialisée,

commission ? La commission partage l'intention des auteurs de l'amendement. Nous considérons que l'importance de cette politique justifierait pleinement la nomination d'un ministre dédié, malgré la grande implication du ministre de l'Europe et des affaires étrangères. Toutefois, cela relève de la décision du Président de la République, sur proposition du Premier ministre.

je vous remercie de vouloir renforcer l'équipe gouvernementale, mais je rejoins

de l'Assemblée nationale, selon laquelle le ministre chargé du développement est compétent pour définir et mettre en oeuvre le politique de développement, en lien avec le ministre de l'économie et des finances.

commission ? Le présent amendement tend à revenir sur des modifications opérées par la commission pour renforcer le rôle du ministre chargé du développement, et ainsi améliorer le pilotage de la politique de développement solidaire. Rappelons que l'alinéa 113, visé par la première partie de l'amendement, mentionne déjà que le ministre chargé du développement « veille avec les ministres chargés de l'économie et du budget et les autres ministres concernés, à la cohérence des positions et de l'affectation des contributions françaises vers les fonds et programmes multilatéraux, et à leur adéquation vis-à-vis des priorités de l'action extérieure de la France Le rôle du ministre chargé de l'économie et du budget est ainsi souligné, dans le champ d'action qui lui est propre. Néanmoins, il semble normal de réaffirmer que la politique de développement solidaire est pilotée principalement par le ministre chargé du développement. Il en va de même du Cicid : cette instance est interministérielle par nature, mais le secrétariat devrait logiquement en être assuré par le principal pilote de cette politique, le ministre chargé du développement solidaire. Nous souhaiterions d'ailleurs,

chaque année, les ministres de tutelle de l'AFD- le ministre chargé du développement et le ministre chargé de l'économie -remettent au directeur général de l'Agence une lettre d'objectifs.

qui constitue une redondance sans pour autant empêcher les élus locaux de participer aux conseils locaux du développement. En effet, les élus locaux de l'Hexagone et d'outre-mer sont déjà pris en considération

Cet amendement vise à inclure les groupes d'amitié parlementaire- ils sont 153 à l'Assemblée nationale et 81 au Sénat -dans la politique d'aide publique au développement. En tant qu'observateurs, ils pourront ainsi suivre et éclairer les conseils locaux du développement. Quel est l'avis de l'avis de la commission ? Les groupes interparlementaires d'amitié ont pour mission de développer des relations avec les assemblées parlementaires de pays ou d'ensemble de pays avec lesquels la France entretient des relations officielles. Ils contribuent à renforcer la présence et l'influence politique, politique, économique et culturelle de la France à l'étranger, et à favoriser le développement de la coopération interparlementaire et de la coopération décentralisée. Les présidents de groupes d'amitié développent une véritable expertise et un réseau de relations qui peuvent être utiles dans la réflexion sur l'aide au développement. Cet amendement vise aussi à ce que leur rôle

les parlementaires tant à la mise en oeuvre de ces dispositifs

Le choix du recours au prêt peut accentuer la dette des pays. Or la France, en termes de ratio prêts-dons au sein de son APD, fait partie des trois plus gros « prêteurs », derrière le Japon et la Corée du Sud,

contre 16 % en moyenne pour l'ensemble des pays du Comité d'aide au développement (CAD) de l'OCDE. De plus, selon la septième revue par les pairs de l'OCDE publiée en juin 2018, au cours de la période 2012-2016,

Par conséquent, la réduction des prêts dans l'aide française doit être une priorité, afin de lutter contre les inégalités mondiales. C'est pourquoi il est proposé que, d'ici à 2025, la part d'APD en dons représente 85 % de l'APD totale.

au plus près des populations, à la fois, pour choisir des projets en cohérence avec les besoins du terrain et pour emporter davantage l'adhésion des populations locales. Nous pourrions ainsi nous inspirer du programme Star 2022 et de son

En effet, au regard de leur situation géographique, ces collectivités constituent de véritables ponts entre la France et le monde. De ce fait, elles contribuent activement à cette politique de développement solidaire et de lutte contre les inégalités. Avec le soutien Avec le soutien de l'AFD et d'Expertise France, elles conduisent des projets de coopération avec les pays qui composent leur bassin régional, par exemple entre la Guyane et le Suriname. a adopté la stratégie Trois Océans, autour des territoires ultramarins et des États voisins dans l'Atlantique, l'Indien et le Pacifique, dans le but d'apporter une réponse globale à des problématiques transfrontalières et une solidarité internationale au service du développement des États voisins des outre-mer. Depuis 2018, ce sont 255 projets qui ont été financés. Aujourd'hui, Expertise France appuie les efforts nationaux de développement humain durable des pays et territoires d'outre-mer (PTOM) des Caraïbes, le Programme en faveur de la résilience, des énergies durables et de la biodiversité marine dans ces PTOM, à hauteur

commission ? Il paraît effectivement utile de mettre davantage en valeur, dans ce projet de loi, les projets de développement menés par les collectivités d'outre-mer dans leurs bassins régionaux. Nous émettons un avis favorable

: « Si des progrès ont été accomplis, les principaux défis restent les mêmes : les flux financiers illicites, l'érosion de la base d'imposition et les pratiques de transfert des bénéfices demeurent une menace permanente pour les assiettes fiscales africaines. Le ratio impôts-PIB des pays africains reste très inférieur à celui des autres régions du monde. Des progrès doivent donc être réalisés en ce qui concerne l'échange d'informations, les négociations de traités et l'utilisation de procédures d'assistance mutuelle pour lutter contre le non-respect, entre autres.

met lui aussi désormais en avant la nécessité d'augmenter les recettes fiscales, par des mesures adéquates. L'ensemble des mesures qui pourraient être prises doivent donc être soutenues, en lien avec les administrations fiscales.

femmes. Sans vouloir réécrire l'histoire, monsieur le ministre, cet amendement vise simplement à remplacer les termes « droits de l'Homme » par ceux de « droits humains », afin que l'ensemble des personnes composant notre planète soient représentées.

il s'agit de la comptabilisation des instruments du secteur privé (ISP). En 2017, l'AFD déclarait : « Pour démontrer sa volonté de construire des ponts entre public et privé, l'AFD compte doubler ses financements alloués au secteur privé d'ici 2020. Avec comme objectif d'atteindre le cap de 50 % de ses financements vers des acteurs dits " non souverains " qui incluent plus globalement collectivités territoriales, ONG, banques, fonds d'investissement et entreprises publiques ou privées. Elle ajoutait : « Une spécificité unique parmi les bailleurs internationaux. » C'est précisément cette spécificité unique que nous mettons car la comptabilisation des ISP en APD se fait au détriment de la part des services sociaux de base dans les pays les plus pauvres. Or c'est au contraire vers ces derniers que nous voudrions renforcer notre effort. Alors que les financements de l'AFD vers le secteur privé ont progressé de 14 à 19 % entre 2016 et 2017, la proportion des financements pour la santé et l'éducation a reculé durant la même période. Il faut inverser la Nous ne mettons pas en cause l'existence de relations commerciales mutuellement avantageuses impliquant le secteur privé- bien au contraire

Je comprends les préoccupations de Pierre Laurent, mais j'ai déjà eu l'occasion de m'exprimer sur les règles définies par le Comité d'aide au développement de l'OCDE.

J'ajoute que cette récente prise en compte des ISP dans la comptabilisation de l'APD française n'a pas conduit à un délaissement de nos autres priorités de développement. La baisse des proportions des financements pour la santé et l'éducation s'explique par une augmentation du volume de l'activité de l'Agence, alors que ces deux secteurs sont d'abord portés par l'activité en subventions. Au reste, la modification unilatérale

Mme Raymonde Poncet Monge. Une aide publique au développement cohérente, performante et efficace dépend aussi de la production de données concernant les populations visées par les différents projets que nous finançons. C'est la collecte des données et leur analyse qui permettent, pour toutes les institutions et les acteurs impliqués, de définir les politiques publiques efficientes et adaptées aux besoins.

empêche de mesurer les résultats d'une politique publique efficace, notamment envers les filles et les enfants. C'est pourquoi nous proposons d'ajouter l'âge afin d'obtenir des données désagrégées par âge et par sexe, ainsi qu'une prise en compte systématique de l'âge dans les indicateurs de résultats. Cela permettrait de rendre visibles les enjeux liés à la fois au genre et à l'âge, donc de définir des politiques publiques plus adaptées. La prise en compte de l'âge permettra également de contribuer à la protection de centaines de millions d'enfants

l'importance de notre amendement est double. Il s'agit, d'une part, d'orienter efficacement et de manière pertinente les politiques publiques, et, d'autre part, de participer à la protection des enfants, des jeunes et des filles en particulier.

Mieux évaluer, c'est permettre une vision au plus près de la réalité de terrain, et donc adapter notre politique en fonction des besoins réels. Cet amendement vise donc à la mise en place d'indicateurs plus précis. Quel est l'avis de

amendement vise à rétablir une disposition qui était prévue dans la loi de finances pour 2017, laquelle prévoyait l'élargissement de l'assiette de la TTF aux transactions intrajournalières. À l'époque, on chiffrait entre 2 et 4 milliards d'euros annuels le rendement estimé de cette mesure, prévue par la directive européenne sur une TTF continentale

Mme Raymonde Poncet Monge. Cet amendement vise à inscrire dans le corps de la loi le devoir de vigilance des acteurs français exerçant une influence à l'étranger, et à y associer les mécanismes qui permettent d'assurer son efficacité. Ce devoir fait partie intégrante de la responsabilité sociétale des acteurs publics et privés français. Il a d'ailleurs été inscrit comme tel dans le CPG. Rappelons également que, afin d'assurer la cohérence de notre action de notre action de coopération internationale, ce devoir concerne l'ensemble des acteurs français publics et privés ayant une influence à l'étranger. L'importance d'appliquer cette obligation au secteur privé était encore soutenue par le secrétaire d'État Jean-Baptiste Lemoyne le 18 février 2020

Casino, pour son rôle dans la déforestation en Amazonie ; Total, dans plusieurs affaires. La survenance encore trop fréquente de ces affaires prouve que nous devons modifier la loi afin d'accompagner nos entreprises à l'étranger dans le changement de leurs pratiques. Nous proposons d'inscrire dans la loi l'obligation pour ces acteurs de prévenir les atteintes graves, mais aussi de faciliter l'identification de ces atteintes par les autorités judiciaires compétentes et la réparation des préjudices qui ont découlé du manquement à l'obligation de vigilance. Les organisations sur l'extrême difficulté que rencontrent les organisations de la société civile, dont les moyens sont limités, pour réunir les éléments nécessaires à la démonstration de la responsabilité de ces acteurs. Pour remédier à cette faiblesse dans la prévention des atteintes, nous proposons le mécanisme suivant : une personne morale qui ne démontre pas avoir pris toutes les mesures nécessaires et en son pouvoir afin de prévenir une atteinte grave est présumée responsable et, par conséquent, obligée de réparer le préjudice que l'exécution de sa vigilance aurait permis d'éviter. Pour ces organismes, dont les services juridiques et les moyens financiers sont largement supérieurs à ceux des organisations de la société civile, ce mécanisme ne représenterait pas une charge lourde et permettrait une mise en oeuvre efficace

est à M. Pierre Laurent. Cet amendement va exactement dans le même sens : il tend à inscrire une obligation de vigilance pour tous les acteurs intervenant dans le domaine de l'aide publique au développement.

souvent visées dans leurs activités de soutien à l'exportation, qui encouragent des modèles contraires aux objectifs centraux de l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), parce qu'elles desservent des modèles agricoles

relatifs au devoir de vigilance. Nous affirmerions ainsi totalement et clairement la volonté de la France d'exiger de nos entreprises un comportement éthique.

ayant connaissance d'atteintes graves envers les droits humains et les libertés fondamentales, de mise en danger de la santé et de la sécurité des personnes ou de l'environnement, Ce mécanisme s'inscrit dans l'approche de notre politique de développement, guidée par le principe de ne pas nuire. Comme l'a souligné le secrétaire d'État Jean-Baptiste Lemoyne lors de la session extraordinaire et environnemental (CESE), il serait impensable que l'État, ses administrations et ses opérateurs ne respectent pas la loi de 2017 relative au devoir de vigilance. Pour autant,

En outre, une législation européenne relative au devoir de vigilance est en ce moment même à l'étude. Le commissaire européen à la justice doit publier un projet de directive au mois de juin prochain. En élèves modèles, prenons un peu d'avance sur cet agenda de travail. de travail. Afin que notre influence à l'étranger ne souffre pas de telles pratiques, et alors même que nous défendons au travers de ce texte le respect et la promotion des droits fondamentaux, je vous demande de voter cet amendement.

du devoir de vigilance des entités privées et publiques, qu'il s'agisse d'atteintes aux droits de l'homme, à la santé, à la sécurité ou à l'environnement. Dans le cadre de sa politique de développement, la France prend en compte l'exigence de la responsabilité sociétale des acteurs publics et privés, qu'elle promeut auprès des pays partenaires et des autres bailleurs de fonds en s'appuyant sur la loi du 27 mars 2017 relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d'ordre.

que la grande majorité des aides concernées sont versées à des organismes publics souverains ou non souverains, et non à des sociétés. Par ailleurs, de nombreuses petites entreprises des pays en développement, qui participent à la mise en oeuvre

Je l'ai déjà souligné, et Mme Carlotti doit le savoir, nous nous appuyons sur la loi du 27 mars 2017 relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d'ordre. L'AFD, qui met en oeuvre l'ensemble de ces mesures, dispose d'ores et déjà d'une liste d'exclusion interdisant tout financement à d'éventuels bénéficiaires susceptibles de poser des risques, dans un très grand nombre de domaines- travail des enfants, commerce des produits illégaux, destruction d'habitats critiques ... Cet engagement de la France à faire en sorte que les investissements privés soient compatibles avec les ODD

M. Richard Yung. Cet amendement vise à rétablir la cohérence entre la politique de développement solidaire et la politique sociale que la France peut mener dans un certain nombre de pays. Quel

Cet ajout semble indispensable, car la ratification de la Convention des droits de l'enfant implique non seulement une action extérieure de la France conforme aux droits de l'enfant et visant leur effectivité, mais également l'application des droits de l'enfant sur le territoire français. Il est donc indispensable que ces droits fassent l'objet d'un suivi au regard de la cohérence des politiques publiques. L'amendement n°

sur les pays prioritaires de notre APD.

Toutefois, il nous paraît utile de les intégrer dans le champ du rapport annuel afin de voir comment ils évoluent.

est en cohérence avec l'engagement de la France d'adhérer au groupe de travail pour l'agenda sur l'identité juridique, et de contribuer au fonds pour l'enregistrement des naissances qui lui est attaché. En effet, il s'agit du seul fonds ayant pour objectif de mener des actions concrètes en vue de l'établissement systématique d'un état civil. Comme l'a rappelé ma collègue Marie-Arlette Carlotti lors de la discussion générale, l'enregistrement des naissances et l'aide à la constitution d'un état civil fiable est fondamental pour que chaque personne soit reconnue et dispose de tous ses droits, et ce tout au long de sa vie.

et le PNUD. Pérennisé en 2019 afin de mettre en place la feuille de route des Nations unies pour l'identité légale pour la période 2020-2030, il doit aider les pays membres de l'ONU en difficulté à atteindre les ODD 16.9 et 17.19 d'ici à 2030 au travers d'actions concrètes. Ainsi, treize pays ont été identifiés pour y mener potentiellement des actions de renforcement de l'état civil.

il apparaît aujourd'hui indispensable que la France apporte une contribution volontaire à ce fonds en faveur de l'enregistrement des naissances et de la délivrance d'actes de naissance. Cet amendement est également l'occasion de proposer à la France d'adhérer à ce groupe et de contribuer à ce fonds afin de donner une forme concrète à son engagement. C'est la raison pour laquelle le rapport au Parlement sur les choix opérés par la France dans l'allocation de ses contributions aux fonds et programmes multilatéraux doit intégrer l'enregistrement des naissances

des années, nous intervenons en appui de tous les pays partenaires sur ce sujet. Nous finançons les organisations internationales spécialisées dans le cadre de l'agenda sur l'identité juridique de l'ONU, que vous avez cité.

Cet amendement rédactionnel part du constat que le terme « concitoyens » est trop restrictif. Nous estimons que la perception des ressortissants étrangers établis sur notre territoire, en particulier les membres des diasporas, doit également être prise en considération, ce que permet le terme « population ». Comme le précise le CPG, les diasporas jouent un rôle essentiel dans le déploiement de la politique de développement solidaire et de lutte contre les inégalités mondiales de la France, du point de vue tant financier que des compétences qu'elles peuvent mettre à disposition de leur pays d'origine.

est ainsi libellé : La parole est à Mme Hélène Conway-Mouret. Nous ne devons pas perdre de vue que les populations des pays partenaires sont les premières destinataires de notre politique d'aide publique au développement. Malheureusement, le plus souvent, ces populations ne perçoivent pas les effets de nos actions, encore moins leur pertinence et leur portée, du fait de l'insuffisance de notre communication à leur égard. Pire encore, notre présence et nos actions au sein des pays en développement, des espaces de plus en plus concurrentiels, font l'objet d'une hostilité qui alimente des discours antifrançais. Le cas du Sahel en est une illustration éloquente. Notre ambassadeur en République centrafricaine, voilà quelques heures, vient de nous le confirmer. Cette ignorance, voire cette hostilité, devrait nous inviter à repenser notre stratégie de communication. Tel est justement l'objet de cet amendement, qui vise à élargir l'évaluation de la perception de notre politique d'aide au développement, non seulement par nos concitoyens mais également par les populations des pays partenaires. Cet élargissement permettrait d'emporter davantage leur adhésion, d'autant que les gouvernants et les élites de ces pays ne communiquent pas forcément sur les projets portés et financés par notre APD. Par ailleurs, il rendrait plus perceptible notre volonté d'accompagner les États destinataires dans la mise en oeuvre de leur politique de développement vers des résultats probants et concrets.

pour l'année 2019, soit 55,2 % de l'aide apportée au niveau mondial. En 2017, un nouveau consensus européen pour le développement a été défini, afin de constituer un cadre commun global pour la coopération européenne. Au sein de celui-ci, l'Union et les États membres s'engagent à avoir une approche globale, à la fois dans la conception du développement et dans les moyens mis en oeuvre. J'ajoute que notre principal opérateur, l'AFD, met en oeuvre des fonds délégués dans le cadre d'opérations financées par l'Union européenne,

l'espoir d'atteindre les ODD d'ici à 2030. Depuis 2018, ce sont plus de 450 de ces contrats qui ont été signés, avec pour principales conséquences une augmentation de l'inégalité d'accès aux services publics, des scandales de surfacturation et, d'une manière générale, un gouffre financier pour les États. Ainsi, ce sont les secteurs stratégiques des infrastructures routières et de transport en général, des services énergétiques ou des services publics de première nécessité qui ont été investis par les grands groupes au travers de ces PPP, avec des concessions s'étalant sur plusieurs décennies. Les résultats sont inquiétants. Le cofondateur du Forum anti-privatisation (APF), le socialiste sud-africain Trevor Ngwane, a résumé en quelques mots la situation : les PPP justifieront une nouvelle vague de privatisations.

plus de 250 millions de dollars pour du gaz inutilisé dans le cadre du projet gazier de Sankofa, l'entreprise concessionnaire n'ayant pas rempli sa part du marché en termes de délais et ayant surévalué les besoins en gaz. Au Sénégal, c'est l'Autoroute de l'Avenir qui a conduit Dakar à contractualiser avec Eiffage. Au bout du compte, l'entreprise a investi 70 milliards de francs CFA, soit quatre fois moins que l'État. Toutefois, en termes de retombées, c'est exactement l'inverse, puisque l'État n'empochera que la TVA et devra en sus rembourser 200 milliards de francs CFA, autant de revenus qui ne seront pas reversés au nécessaire développement des services nationaux. Pour toutes ces raisons, le recours problématique aux PPP nécessite, à notre avis, d'être mis en lumière. L'APD française ne doit pas s'engager dans le soutien à cette voie. Jean-Marc Todeschini. Cet amendement le souligne, l'un des objectifs de ce projet de loi est de veiller à inscrire l'aide au développement dans un cadre de transparence et de redevabilité exigeant. Une part de plus en plus importante de l'APD et des soutiens publics français destinés au secteur privé vers les pays en développement est opérée des fonds d'investissement, parfois localisés dans des territoires opaques ou à fiscalité faible. La publication de l'intégralité des engagements financiers des agences de l'État et de leurs filiales, ainsi que la mention des intermédiaires financiers et bénéficiaires finaux de ces engagements, permettra une réelle traçabilité et redevabilité de ces actions. Les bénéficiaires finaux sont trop rarement connus quand les opérateurs ont recours à des intermédiaires financiers, ce qui ne permet pas de s'assurer de la destination finale des soutiens. Cette publication permettra également de s'assurer que ces intermédiaires financiers ne sont pas localisés dans des territoires opaques, dans une démarche d'évitement de l'impôt. Alors que le nombre de PPP augmente, la publication de ces contrats et des passations de marchés doit permettre d'entamer une démarche de transparence, en France et dans les pays concernés. ? Mon argumentaire vaudra pour les deux amendements. Il reviendra à la commission indépendante d'évaluation, que nous évoquerons lors de l'examen de l'article 9, de contribuer à la redevabilité et à la transparence de la politique de développement solidaire. Le rapport au Parlement prévu à l'article 2 n'a pas vocation

de l'intégralité des activités opérationnelles du groupe, selon les standards internationaux, à la fois les directives de l'OCDE et les normes de l'Initiative internationale pour la transparence de l'aide (IITA). La politique de transparence de l'AFD prévoit également la publication d'un grand nombre de documents : politiques internes, stratégies d'intervention, rapports financiers semestriels, rapports d'activité et de responsabilité environnementale et sociale, et comptes

L'ajout que nous proposons semble indispensable, car la ratification de la Convention internationale des droits de l'enfant implique une action extérieure de la France conforme aux droits de l'enfant et visant leur effectivité. L'ONU rappelait en mars dernier qu'en 2020, à la suite de la pandémie, le nombre d'enfants vivant dans la pauvreté avait augmenté de 142 millions. Ce chiffre s'ajoute à celui des 663 millions d'enfants qui vivaient déjà dans la pauvreté, selon l'Unicef. Des dizaines de millions d'enfants ont été déscolarisés, des dizaines de millions d'autres ont perdu un parent, voire les deux, et se retrouvent en situation d'extrême vulnérabilité. 172 millions d'enfants sont encore victimes de travail forcé, 5 millions d'enfants de moins de cinq ans meurent encore chaque année de maladies, de faim et de maltraitances dues à la pauvreté. Les droits de l'enfant doivent être visibilisés. Il s'agit non pas d'un ajout esthétique ou d'une précision superflue, mais de la protection des enfants et des engagements de la France dans le cadre de la Convention internationale des droits de l'enfant, de sa responsabilité en tant que pays donateur d'orienter ses politiques publiques dans un cadre législatif clair prenant en compte les plus vulnérables, dont les enfants.

d'ailleurs l'occasion qui m'est donnée pour apporter tout le soutien de notre groupe aux acteurs de terrain, et pour saluer l'engagement des militaires de l'opération Barkhane et celui des acteurs du développement au Sahel. La pression militaire permanente a permis d'éviter la constitution d'un sanctuaire djihadiste. Comme chacun le sait, la solution devra aussi être politique, économique et sociale. Elle impliquera un volet « reconstruction », dans lequel l'action des acteurs du développement sera déterminante. Je salue le rôle joué par la coopération décentralisée et les jumelages entre nos communes françaises et celles du Sahel. On peut citer à cet égard la ville d'Orsay et la commune nigérienne de Dogondoutchi, ou la Bretagne et le nord de Madagascar.

nous avons besoin d'une plus grande transparence. La doctrine consistant à combiner la défense, la diplomatie et le développement, appelés les « 3D », n'est pas forcément très équilibrée. Il suffit de parcourir le rapport de la Cour des comptes sur les actions civiles et militaires de la France dans les pays du G5 Sahel, publié le 22 avril 2021, pour comprendre très vite que la majorité des sommes

pays de la bande sahélo-saharienne est parfois remise en cause et fait l'objet d'un certain ressentiment de la part de populations qui peinent à voir, dans leur vie quotidienne, les résultats du développement promis. Il est donc important et urgent que notre action s'inscrive à l'aune du contexte politique, et surtout social, de ces pays. La politique étrangère de la France est déterminante, tant pour la sécurité et le développement socio-économique du Sahel que pour notre sécurité, dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Les complémentarités entre actions militaire et civile d'aide à la stabilisation et au développement fait, à parité les moyens que nous devons consacrer au développement. Cet amendement vise donc à offrir une meilleure grille de lecture de nos efforts en faveur du développement, en veillant, dans la présentation de la distribution des ressources, à ce que la dimension « développement » soit une composante à part entière de la politique étrangère de la France à l'égard des pays partenaires. Il s'agit également de contribuer au renforcement du droit de regard du Parlement sur la répartition des ressources affectées aux 3 D. Quel est l'avis de

Ce rôle essentiel est reconnu par le Gouvernement qui, dans ce texte, se donne les moyens de promouvoir l'accès de toutes et de tous au dispositif de volontariat à l'international et de développer des volontariats

L'article 48 de la Constitution prévoit que l'ordre du jour est fixé par chaque assemblée. Il ne revient pas à une disposition d'une loi de programmation de contraindre l'ordre du jour des assemblées parlementaires. Une telle disposition ne nous paraît donc pas nécessaire. Quel est l'avis de

collègue soit exact : cette disposition n'est absolument pas nécessaire pour qu'un débat parlementaire annuel ait lieu. Pour autant, nous considérons qu'elle a une valeur politique et symbolique et qu'elle conforte le rôle du Parlement dans le contrôle de la politique d'APD. Il nous paraît

trop déclarative et assez peu contraignante, y compris sur la question du droit d'initiative. C'est pourquoi les membres de la commission ont voulu, à la quasi-unanimité, consacrer un article à la société civile, en affirmant la dimension partenariale. Pour le Sénat, les associations sont non pas de simples prestataires, mais de réels partenaires, tant dans l'élaboration que dans la mise en oeuvre de la politique de développement. Les associations qui ont suivi nos travaux se sont réjouies de la position des sénateurs et de cet article spécifique, dans lequel elles se reconnaissent et qu'elles réclament depuis longtemps. Le CESE, dans un avis de février 2020, préconisait

pouvait transformer l'alinéa 8 de l'article 1 en un article complet dédié à la société civile ». C'est ce que nous avons fait ! Je pense donc que le Gouvernement soutiendra cette proposition, et je souhaite que M. Yung retire les amendements qu'il

Néanmoins, notre devoir étant de nous assurer que ce que nous votons est clair et lisible, nous proposons de remédier à une redondance rédactionnelle entre les alinéas

En effet, le premier alinéa revient à souligner le rôle essentiel joué par ces acteurs, tandis que le deuxième appelle l'État à les associer au déploiement de la politique de développement solidaire. Nous souhaitons donc, à des fins de clarification de cet

justement pour objet les volontariats réciproques. C'est parce que l'État reconnaît leur effet de levier transversal qu'une disposition entière est consacrée au développement et au régime juridique de ces volontariats. que nous venons de voter un amendement du groupe RDPI, qui intègre dans le champ du rapport annuel transmis au Parlement le bilan des actions menées par le Gouvernement

qui a justement pour objet les volontariats réciproques. C'est parce que l'État reconnaît leur effet de levier transversal qu'une disposition entière est consacrée au développement et au régime juridique de ces volontariats. Je rappelle également que nous venons de voter un amendement du groupe RDPI, qui intègre dans le champ du rapport annuel transmis au Parlement le bilan des actions menées par le Gouvernement en matière de volontariats réciproques. Quant au rapport annexé, il dispose également, à l'alinéa 23, que « La France encourage l'accès de tous, en veillant à intégrer celles et ceux qui vivent en situation de pauvreté ou de vulnérabilité, aux dispositifs dispositifs de volontariat à l'international, y compris dans le cadre de la mobilité croisée et des volontariats réciproques ». Il n'apparaît donc pas utile de le préciser à nouveau dans cet article 2 .

qui reconnaît le rôle des différents partenaires et promeut le volontariat. Or cet alinéa est indissociable du suivant, qui fixe le principe d'association des OSC dans le cadre d'un dialogue annuel. Avis défavorable,

vise à supprimer la référence au volontariat dans cet article qui consacre le rôle des OSC, mais aussi des citoyens, dans la politique de développement solidaire. La référence au volontariat a pourtant toute sa place dans un alinéa qui consacre le rôle de la société civile. Avis défavorable.

de la commission ? La question du droit d'initiative des OSC a été traitée à l'article 1, qui prévoit un dispositif dédié pour les projets présentés par les OSC.

L'ordonnance n° 2020-1342 du 4 novembre 2020 qui a procédé à cette transposition et qui renforce l'application des mesures de gel des avoirs et d'interdiction de mise à disposition a en effet occulté son application aux organisations de solidarité internationale, et fait potentiellement obstacle à la mise en oeuvre de l'action humanitaire par ces organisations. Dans les faits, seraient ainsi sanctionnées désormais la simple mise à disposition ou l'utilisation de fonds et ressources économiques au profit de certaines personnes, ce qui concernera les soins et les vivres, y compris à l'étranger, sans que soit prévu le caractère intentionnel ou non de l'infraction supposée. En tant qu'elle ne prévoit aucune exemption humanitaire, cette ordonnance aurait pour effet de remettre en cause les conditions et principes d'intervention des organisations humanitaires et de solidarité internationale, de criminaliser les activités relevant de l'action humanitaire et de faire peser sur les organisations de solidarité présentes sur le terrain le risque de poursuites et de condamnations pénales. Cette ordonnance aurait déjà des répercussions sur la poursuite même des activités sur le terrain. Dans l'attente d'une mise en conformité avec les obligations découlant de cette ordonnance et d'une clarification du droit applicable, certains bailleurs de fonds chargés de procéder au criblage des bénéficiaires finaux, comme l'AFD, ont suspendu des contrats de financement, provoquant le blocage des opérations concernées par ces contrats.

nécessaire prise en compte des organismes à but non lucratif dans l'édiction de mesures de lutte contre le financement du terrorisme, selon une approche fondée sur les risques et sur des mesures ciblées et proportionnées. la directive du 15 mars 2017 relative à la lutte contre le terrorisme, pierre angulaire du cadre juridique de l'Union européenne en la matière, exclut bien de son champ d'application les activités humanitaires.

de mon point de vue, nous ne visions que les actions humanitaires et les associations humanitaires. Peut-être est-il mal rédigé ; en conséquence, et à ce stade, tout en vous disant que nous ne faisons pas preuve de laxisme, nous allons retirer cet amendement.

pour tout le monde.

au détriment, par exemple, de l'accord de Paris. Nous proposons de maintenir telle quelle la première phrase de l'article L. 115-1 du code général des collectivités territoriales, qui fixe le principe et le cadre général de l'action extérieure des collectivités territoriales et la répartition des compétences avec l'État, et de déplacer cette mention de l'Agenda

Rappelons-le : ces dispositifs nés en 2005 avec la loi Oudin-Santini permettent d'attribuer aux collectivités des ressources propres pour le financement du développement solidaire dans les secteurs de l'eau, de l'énergie et du traitement des déchets. Dans ce contexte, il nous semble particulièrement utile de faire une de ces dispositifs, alors que la place des collectivités territoriales est mise en valeur dans ce texte. Pour rappel, ce sont environ 5 000 collectivités territoriales qui mènent aujourd'hui des actions de coopération avec des collectivités étrangères. L'aide publique provenant des collectivités locales représente 2,6 % de l'APD totale, une proportion relativement élevée en comparaison avec les autres pays du Comité d'aide au développement. Toutefois, selon le rapport du député Hervé Berville, seul le dispositif « 1 % eau et assainissement » est aujourd'hui réellement utilisé, sachant que presque 10 % de l'APD des collectivités proviennent des syndicats franciliens des eaux et de l'assainissement.

commission ? Un point très complet est déjà effectué chaque année dans le cadre du rapport sur l'aide publique au développement des collectivités territoriales réalisé sous l'égide de la CNCD.

? Mon administration est en mesure de préparer un rapport spécifique sur la mise en oeuvre et les résultats de l'action extérieure des collectivités territoriales les dispositifs

ainsi adopté a eu pour effet de supprimer la mention de la possibilité d'effectuer des missions d'intérêt général. Aujourd'hui, devant la multiplication des catastrophes climatiques, des crises humanitaires et des conflits, une telle suppression paraît injustifiée. Les acteurs humanitaires et ceux du développement ne sont pas exactement les mêmes. Le présent amendement vise donc à remédier à cette suppression.

à la politique publique de développement veillent à ce que les projets qu'ils soutiennent ne participent pas à la privatisation des services publics dans les pays récipiendaires. Les exemples sont nombreux d'efforts publics ou de soutiens à des

en rend l'accès totalement impossible à la grande majorité de la population, ce qui est évidemment contraire à l'objectif de l'APD. Il nous paraît donc important de préciser cet objectif de non-privatisation des projets publics que nous soutenons l'APD.

beaucoup de nos collègues ont eu l'occasion de dénoncer un certain nombre d'errements, comme je les qualifie volontiers, et en tout cas de s'étonner que la politique publique de développement de la France se fasse, par exemple, en direction de la Chine ou de la Turquie au moment où celles-ci fustigeaient le Président de la République. La Cour des comptes s'est également émue de quelques difficultés de fonctionnement. À étudier les données budgétaires

ce qui, dans le contexte budgétaire que nous connaissons, appelle à une certaine vigilance. On demande à l'ensemble des administrations de l'État de

politique et stratégique d'une administration sous tutelle du ministère de l'économie et des finances et du ministère des affaires étrangères. Cela est d'autant plus indispensable que les crédits gérés par l'AFD atteignent les 14 milliards d'euros. Par ailleurs, et à l'issue de ce parcours législatif, l'AFD fonctionnera comme une véritable holding, avec ses filiales Proparco et Expertise France. L'AFD va ainsi devenir le fer de lance de l'aide publique française. Par conséquent, la redéfinition de ses missions, leur hiérarchisation et leur ciblage géographique sont indispensables. De même, il est impératif que l'Agence soit exemplaire et fasse preuve de davantage de transparence, tant sur le volet financier, notamment dans ses prises de participation financière dans les autres banques de développement, qu'en matière de publication précise de tous les projets qu'elle finance. La traçabilité des fonds et des activités doit être exigée. Il importe enfin qu'une vigilance accrue soit de mise, alors que le seuil critique d'endettement de nombreux pays africains auxquels elle alloue des prêts est atteint. Selon le FMI, sur les dix-neuf pays prioritaires de l'aide française, sont en situation de risque modéré ou élevé. Il semble ubuesque que les fonctionnaires de Bercy n'appliquent pas la doctrine Lagarde interdisant l'allocation de prêts souverains aux pays considérés comme à risque de surendettement

à la volonté des sénateurs de distinguer la mission de l'agence dans les pays les moins avancés (PMA), en particulier dans les pays prioritaires, de celle qui vise à financer les biens publics mondiaux, dont le climat, dans l'ensemble des pays en développement. Nous souhaitons renforcer encore cette disposition

de la commission nous conforte dans cette direction ! Il me paraît par ailleurs important de ne pas formuler les missions de l'AFD de manière trop prescriptive afin de préserver la capacité de l'Agence à intervenir aussi dans les PMA dans les domaines de la gouvernance, de la stabilisation ou encore du climat et de l'environnement, ainsi que sous forme de garanties et de prises de participation dans ces pays. Nous ne souhaitons pas, en effet, priver les pays prioritaires des actions que pourront mener nos opérateurs dans ces domaines en particulier, qui ne sont pas réservés aux pays à revenu intermédiaire ou émergents. Il est enfin important de préserver la capacité de l'AFD à financer l'accès aux services essentiels de l'ensemble des pays en développement, y compris dans les pays à revenu intermédiaire, dans le contexte sanitaire que nous connaissons. Cet amendement vise à enrichir

ou alors très peu. Il me paraît donc légitime que l'on puisse tenir compte de cette situation. J'ai eu l'occasion, dans un autre cadre, de rédiger un rapport sur la situation de l'île de la Passion-Clipperton.

Laurent. Cet amendement vise à assurer le pluralisme de la représentation parlementaire au sein du conseil d'administration de l'AFD.

Nous nous réjouissons que la France ait adopté le qualificatif de diplomatie « féministe », bien que cela reste encore un objectif de notre politique et ne soit pas tout à fait une réalité effective. Afin que l'ensemble de la politique de développement de la France se mette en cohérence avec ses ambitions féministes, nous souhaitons inscrire dans cet article la nécessité que les parlementaires

de l'AFD tend à le montrer. La récente désignation tant de Mme Isabelle Briquet que de M. Alain Joyandet comme représentants de la Haute Assemblée prouve que chacun accorde de l'importance à cette parité et qu'elle est bien effective à chaque nomination.

la présence de représentants des ministères compétents de l'aide publique au développement, en particulier du ministère chargé de l'écologie, qui est le seul ministère parmi ceux qui sont mentionnés à ne pas avoir encore de représentants au sein de ce conseil. Sa représentation est pourtant essentielle si l'on souhaite réellement mettre en oeuvre, en coordination avec les autres ministères compétents, la réalisation de l'Agenda 2030.

à la définition de la lettre d'objectifs adressée au directeur général de l'AFD, conformément à un souhait de notre assemblée. Compte tenu de l'importance prise par le développement durable dans les objectifs de l'AFD, qui s'est engagée à devenir 100 % compatible avec l'accord de Paris, un tel ajout semble pertinent.

L'intégration de la société Expertise France au sein de l'Agence française de développement est saluée par beaucoup comme un gage supplémentaire de la qualité de notre action de coopération, en dotant l'AFD d'une composante « expertise », essentielle pour l'optimisation de ses capacités ; ensuite, en assurant à Expertise France une pleine participation à la politique d'aide au développement et un volume d'activité accru. Cette intégration est une démarche que nous soutenons, même si nous constatons que, dans les faits, ce rapprochement est déjà largement engagé et que le rôle du Parlement à cet égard relève davantage de la reconnaissance d'un fait accompli que

opérationnelles, logistiques et financières, afin que le processus soit générateur de sens pour les salariés des deux opérateurs. Parmi ces opportunités, l'étude d'impact fait mention de nouvelles perspectives de carrière pour les salariés d'Expertise France.

Expertise France pour bénéficier d'un appui renforcé dans la mise en oeuvre de leur action extérieure. Nous proposons de maintenir la mention explicite aux collectivités territoriales d'outre-mer.

Cet amendement technique vise à préciser la procédure de nomination de l'administrateur représentant les organisations de la société civile et de l'administrateur représentant élu des collectivités territoriales. Nous proposons une nomination par décret, qui est similaire à la procédure suivie pour la nomination des